L'ordre du jour appelle l'examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l'approbation de conventions internationales. Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure d'examen simplifié. Je vais donc les mettre successivement aux voix. Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole

Je mets aux voix le texte adopté par la commission sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole d'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Macédoine du Nord

signé à Bruxelles le 7 février 2019. Avec l'entrée en vigueur de ce protocole, la Macédoine du Nord deviendra le trentième allié de l'OTAN. Je rappelle que, lors de sa création, en 1949, cette

Depuis vingt ans, la Macédoine du Nord a réalisé des progrès constants pour la mise en oeuvre du MAP : je pense à la réforme des secteurs de la défense et de la sécurité, à l'accroissement de l'interopérabilité au plan militaire, ou encore à la lutte contre la criminalité organisée et la corruption.

Pour la France, l'élargissement de l'OTAN n'est aujourd'hui ni une priorité ni une fin en soi. Il ne peut être envisagé que dans la mesure où il renforce effectivement la sécurité de l'espace euro-atlantique et la crédibilité de la défense collective. il n'existe pas aujourd'hui de consensus quant à l'adhésion de la Bosnie-Herzégovine, dernier candidat dans la région, et, plus à l'est, de l'Ukraine ou de la Géorgie ; et il n'y aura pas de nouvel élargissement s'il n'y a pas de consensus quant à la contribution de nouvelles adhésions à la sécurité de l'espace euro-atlantique.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, c'est la demande de notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées que nous examinons aujourd'hui en séance publique le projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Macédoine du Nord. Un nouvel élargissement de l'OTAN, en effet, n'est pas quelque chose d'anodin. Malheureusement- force est de le souligner -, celui-ci survient à un moment où l'Alliance euro-atlantique est mise à mal par ses divisions et ses contradictions. Face à la crise qui se déroule actuellement dans le nord-est de la Syrie, l'OTAN semble paralysée, incapable de réagir à l'intervention militaire de l'un de ses membres, la Turquie, contre nos alliés dans la lutte contre Daech, les Kurdes. Quant aux États-Unis, ils ont laissé faire la Turquie et ont opté pour le retrait de leurs troupes.

Au terme du processus de ratification, la Macédoine du Nord deviendra le trentième pays de l'Alliance atlantique. Au total, vingt-trois des États membres de l'OTAN, ainsi que la Macédoine du Nord elle-même, ont déjà ratifié le présent protocole. Si tout se passe bien, l'accession de la Macédoine du Nord à l'OTAN sera entérinée lors du prochain sommet de l'OTAN, à Londres, en décembre 2019. J'espère que l'Assemblée nationale se saisira très vite après nous de ce dossier Depuis son indépendance, la Macédoine du Nord a fait le choix résolu de se tourner vers l'OTAN et vers l'Union européenne. Toute la génération née après l'indépendance a grandi dans la promesse et le rêve d'un avenir euro-atlantique. Pourtant, si cet État s'est vu accorder le statut de pays candidat à l'Alliance et le bénéfice du plan d'action pour l'adhésion en 1999, toute avancée est restée longtemps bloquée du fait du litige avec la Grèce sur la fameuse question du nom. en 2008, lors du sommet de l'OTAN organisé à Bucarest, qui a donné le feu vert aux négociations avec l'Albanie et la Croatie, les alliés ont soumis l'ouverture de négociations avec l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, l'ARYM, à la résolution de la question du nom. Après des années de, les négociations entre les deux voisins ont repris en 2017 grâce à une volonté politique des gouvernements grec et macédonien. De manière assez inattendue, elles ont abouti à la signature de l'accord de Prespa le 17 juin 2018. Aux termes de cet accord, l'ARYM a pris le nom de Macédoine du Nord, tant vis-à-vis de l'extérieur qu'au plan intérieur. Cet accord a ouvert au pays la voie de l'accession à l'OTAN. Dès le mois suivant, en juillet 2018, les négociations d'adhésion ont été lancées, aboutissant à la signature du présent protocole le 6 février 2019. Indéniablement, la perspective de l'adhésion à l'OTAN a favorisé les réformes et les progrès en Macédoine du Nord. En attestent les rapports établis chaque année dans le cadre du plan d'action pour l'adhésion renforcement des standards de la police, lutte anticorruption, coopération avec Europol, adoption de documents stratégiques dans le domaine de la défense, renforcement de l'interopérabilité avec les forces de l'OTAN, Bien sûr, la Macédoine du Nord doit encore progresser en matière d'État de droit et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. Néanmoins, s'agissant du dossier otanien, force est d'admettre que, avec la signature de l'accord de Prespa, la Macédoine du Nord a surmonté le principal obstacle qui s'opposait encore à son adhésion. Certes, la contribution financière de la Macédoine du Nord au budget de l'Alliance sera modeste, de l'ordre de 1,7 million d'euros par an. Il en est de même de son budget de la défense, qui s'élève à 101,3 millions d'euros en 2018, soit un peu plus de 1 % du PIB du pays. Il devrait toutefois être augmenté de 0,2 % par an jusqu'en 2024, afin de tendre vers l'objectif des 2 %. Cet effort permettra au pays de moderniser ses forces armées, qui sont pour l'essentiel terrestres, et surtout de renouveler leurs équipements qui sont totalement obsolètes. En outre, la Macédoine du Nord prend part aux opérations extérieures de l'OTAN, avec une contribution de 47 soldats à l'opération en Afghanistan et un soutien logistique de la KFOR au Kosovo. Elle participe également à la mission européenne Althea en Bosnie-Herzégovine et pourrait envoyer prochainement, dans le cadre d'un arrangement bilatéral avec la France, deux officiers au titre de l'opération EUTM RCA, ce qui va dans le sens de nos objectifs en Afrique

appliquée aux pays de l'est de l'Europe après la fin de la guerre froide. Cette démarche est d'abord politique : elle vise à conforter la sécurité des alliés en promouvant la paix, la liberté et la démocratie. Comme l'a dit l'une des personnalités que nous avons auditionnées lors de la préparation de mon rapport, « l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN cimente une dynamique vertueuse d'apaisement des tensions régionales

Certes, les considérations géopolitiques ne sont pas absentes, compte tenu du rôle joué dans la région par des puissances extérieures comme la Russie ou la Chine. Pour autant, la Macédoine du Nord ne ressent pas de menace extérieure particulière. L'adhésion à l'OTAN est avant tout perçue, notamment par sa population, comme le corollaire d'un rapprochement avec l'Union européenne, qui nourrit de fortes aspirations pour des raisons avant tout socio-économiques. En effet, elle porte en elle l'espoir d'un développement économique du pays, massivement touché par l'émigration des jeunes. un mot de la position française quant à cette adhésion. La France se montre traditionnellement prudente, pour ne pas dire réticente, face aux élargissements de l'OTAN : elle a pour préoccupation d'atténuer les malentendus qui pourraient en découler dans ses relations avec la Russie. Pour elle, l'élargissement de l'OTAN ne saurait être une fin en soi, toute candidature à l'adhésion devant être évaluée à l'aune de sa capacité à contribuer à la stabilité de l'Alliance. S'agissant de la Macédoine du Nord, la France était opposée à l'adhésion tant

la conduisent à donner son feu vert. Mes chers collègues, notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a adopté ce projet de loi la semaine dernière.

avec lequel nos relations bilatérales sont tout à fait favorables et dont une grande partie de la société exprime une attirance culturelle vers la France : M. le secrétaire d'État a très judicieusement rappelé

l'esprit qu'il s'agit d'un État bicommunautaire, avec une composante majoritaire slavophone et une minorité albanophone, assez concentrée territorialement et en croissance démographique.

Or, le 10 septembre 2001- la veille du 11 septembre -, nous avons salué un communiqué du département d'État affirmant que les forces européennes de défense seraient les mieux placées pour assurer l'application du cessez-le-feu.

pour commencer, je tiens à remercier le président de la commission, Christian Cambon, d'avoir demandé l'inscription en séance publique de ce débat sur la ratification de la convention d'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN. C'est en effet un sujet d'importance, qui ne saurait être expédié sans réflexion.

dans l'OTAN de tous les pays des Balkans issus de l'éclatement de la Yougoslavie et de la guerre qui a ensanglanté la région. En vérité, les États-Unis ont alors entrepris ce qu'ils appellent encore aujourd'hui « l'extension de la ligne de front de l'OTAN vers la Russie concerne les Balkans et tous les pays de l'est de l'Europe jusqu'à l'Ukraine. En 2003 était signée la charte de l'Adriatique avec les États-Unis, qui poussait les feux de ce projet et constitue jusqu'à aujourd'hui le motif premier de cette adhésion. C'est ce projet américain qui enregistrera un nouveau progrès si nous ratifions aujourd'hui cette adhésion, dont le ressort principal ne relève donc pas d'un projet partagé de sécurité régionale, mais bien de l'accélération du processus d'élargissement de l'OTAN vers l'est de l'Europe, sous impulsion américaine. Il y a presque trois ans, notre chambre débattait de l'adhésion du Monténégro à l'OTAN, intervenue en 2017. Cohérent, notre groupe soulignait déjà dans ce débat les dangers de la militarisation atlantiste de la zone balkanique, qui, loin d'améliorer sa sécurité,

Selon l'Organisation internationale du travail, la pauvreté touche 41 % de la population de Macédoine du Nord. N'y a-t-il pas de priorité

sont les premiers à repousser aux calendes grecques l'intégration économique et politique de ces pays. Dès lors, ils ne peuvent même pas nous expliquer qu'il s'agit de jeter les bases d'un futur de système de défense européen, puisque la Macédoine du Nord adhérera à l'OTAN, mais sera soigneusement maintenue dans l'antichambre de l'Union européenne, sans espoir d'en sortir à court ou à moyen terme. terme. Quel est donc le sens de cette adhésion, qui sonnera comme une victoire pour les États-Unis au moment même où ceux-ci et leurs alliés turcs, également très actifs dans la région balkanique, viennent de provoquer une crise majeure de l'OTAN en tournant le dos à leurs alliés européens de la coalition en Syrie et en lançant une offensive condamnée par nous tous contre les Kurdes ? L'adhésion d'un trentième pays à l'OTAN est dangereusement anachronique. Elle torpille toute velléité d'une réflexion indépendante sur un nouveau système de sécurité collective en Europe. Elle tourne le dos aux autres modèles de coopération nécessaires. Elle affaiblit le rôle de l'ONU au profit d'un système aligné, désuet et dangereusement miné par outrances américaines et par les contradictions entre ses principaux contributeurs.

Comme le rappelle le Président de la République fédérale d'Allemagne : « Celui qui croit augmenter le niveau de la sécurité avec des parades de chars sur le front est de l'alliance se trompe ». Tel est pourtant l'objectif sans cesse énoncé par le secrétaire général de l'alliance atlantique. Il faut cesser d'urgence la course à la confrontation dans laquelle l'OTAN joue un rôle de premier plan, comme le montre son action de plus en plus contestable dans les récentes crises et conflits internationaux et, tout au contraire, relancer d'urgence l'initiative politique pour une nouvelle conférence paneuropéenne sur la sécurité collective du continent. L'OTAN a besoin non pas d'un trentième adhérent, mais de la tenue d'un débat parlementaire en urgence, dans lequel nous, parlementaires français, prendrons le temps d'évaluer le sens de la situation et de cette alliance, ainsi que notre rôle au sein de son commandement intégré. Arrêtons la machine infernale de l'escalade militaire qui s'est remise en route au plan mondial

N'y voyez pas un geste de défiance à l'égard de la Macédoine du Nord : notre vote est un appel à reprendre d'urgence notre destin en main, loin des visées bellicistes dans lesquelles, à défaut, la France et l'Europe risquent de se trouver entraînées

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la Macédoine du Nord est née en 1991 de l'ancienne Yougoslavie. Depuis près de vingt ans, ce pays est un partenaire fiable de l'OTAN, qui participe déjà à certaines opérations, dont en Afghanistan.

Ainsi, la république de Macédoine du Nord est sur le point de devenir le trentième État membre de l'OTAN, une organisation qui a fêté cette année ses soixante-dix ans d'existence et qui continue d'être efficace, comme l'ont montré ses interventions dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak et en Libye. L'OTAN a évolué au cours de son histoire. Conçue dans le contexte de la guerre froide comme un rempart au péril stalinien, elle a perduré après l'effondrement de l'Union soviétique et a été progressivement élargie aux pays d'Europe, à la Turquie et à d'anciennes Républiques du bloc communiste, en 1999 et en 2004. Ces élargissements, issus de la politique dite « de la porte ouverte », ont donné lieu à des tensions avec la Russie, qui voit ces pays s'éloigner un peu plus de sa sphère d'influence.

Pendant longtemps, l'OTAN représentait la promesse d'une protection assurée par les États-Unis. Elle a participé, avec les « dividendes de la paix », évoqués dans les années 1980 par le Premier ministre Laurent Fabius, à la dégradation des capacités de défense des pays européens.

Depuis le sommet de Saint-Malo en 1998, ces deux pays constituent le coeur de la défense européenne. Nous verrons peut-être le Royaume-Uni quitter l'Union à la fin du mois. Cela ne constitue pas une bonne nouvelle, en particulier pour la défense de l'Europe, qui verrait partir l'un de ses deux piliers.

doit nous interpeller, parce que les États-Unis, comme d'autres, pourraient avoir intérêt à conserver une Europe dans un état de dépendance. Or le président américain affirme que les États-Unis ne peuvent plus être le gendarme du monde. Il est à craindre que nos alliés américains portent leurs efforts sur d'autres zones- doctrine Monroe » ou « pivot asiatique » -, au détriment de la protection de nos territoires. Dans ce contexte, l'OTAN ne peut pas reposer sur la seule initiative américaine. Pour perdurer, cette organisation a besoin de nouveaux membres, comme la Macédoine du Nord. Le désinvestissement des États-Unis met aussi en lumière combien il est crucial que les pays européens soient autonomes. L'Europe doit pouvoir assurer sa propre défense afin de faire entendre sa voix, dans l'intérêt de ses membres. À l'heure d'une nouvelle mandature et d'une nouvelle composition des organes dirigeants de l'Union européenne, il faut tendre vers plus d'intégration, ainsi, d'ailleurs, que de plus en plus d'États européens le proclament haut et fort. L'Europe est en crise, notamment idéologique. Elle doit se renouveler pour perdurer. La définition de la politique de défense européenne est incontournable, car elle doit parvenir à une autonomie stratégique. Je veux saluer ici le travail de mes collègues Ronan Le Gleut et Hélène Conway-Mouret, qui ont produit un rapport éclairant sur la défense européenne et le défi de l'autonomie stratégique. Le Président de la République a appelé de ses voeux une meilleure intégration. Cette dynamique est enclenchée. Le Fonds européen de la défense finance déjà des projets communs de recherche dans ce domaine, mais il reste beaucoup à faire pour parvenir à cette autonomie. et territoires votera en faveur de l'accession de la Macédoine à l'OTAN. Nous souhaitons cependant que les élargissements ne fassent pas oublier la nécessité, pour l'Europe, d'atteindre l'autonomie stratégique, ainsi qu'une plus grande intégration de ses moyens de défense.

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons ce matin le projet de loi autorisant la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Macédoine du Nord. du Nord. Depuis 1991, la Grèce a toujours mis son veto à l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN. Athènes s'opposait à ce que cet État, issu de l'éclatement de la République fédérale de Yougoslavie, porte le même nom qu'une de ses régions, la Macédoine. Macédoine. Ce désaccord sur la dénomination de ce petit pays des Balkans a cristallisé bien des passions, de part et d'autre de la frontière, et a toujours été le principal facteur de blocage de son adhésion à l'OTAN, adhésion qui nécessitait l'accord de l'ensemble des membres de l'organisation, donc de la Grèce. Comme cela a été souligné par mes collègues, l'accord de Prespa de juin 2018, signé par Athènes et Skopje, a débloqué la situation pour que, enfin, la Macédoine du Nord puisse entamer son processus d'adhésion. Devenir membre de cette alliance ouvre la voie à l'intégration de ce pays dans la communauté occidentale et constitue un marqueur identitaire fort, mais aussi un symbole de reconnaissance internationale. Cette accession illustre également l'aboutissement de progrès importants réalisés dans le cadre du plan d'action pour l'adhésion. L'intérêt d'accueillir ce trentième membre au sein de l'OTAN ne saute peut-être pas aux yeux, puisque la Macédoine du Nord reste un pays en proie à de nombreuses difficultés et dont les forces armées demeurent modestes. Cependant, son adhésion permettra de renforcer la stabilité des Balkans occidentaux et d'amoindrir les tensions avec la Bulgarie et l'Albanie. La Macédoine est la quatrième des six ex-républiques yougoslaves à adhérer à l'OTAN, après la Slovénie, la Croatie et le Monténégro. Cette démarche s'inscrit avant tout dans la politique dite « de la porte ouverte » visant à encourager la « sécurité coopérative », la paix et la démocratie. Certains y discerneront une éventuelle intention de l'OTAN de réduire l'influence russe dans la région. à ce sujet de rappeler la prudence de la France, qui a pour préoccupation majeure d'atténuer les malentendus qui pourraient découler des élargissements de l'OTAN, dans le cadre des relations avec la Russie. Comme l'a rappelé notre rapporteur Joëlle Garriaud-Maylam dans son rapport, notre pays a à coeur de soutenir que toute candidature doit, avant tout, être évaluée en fonction de sa capacité à contribuer à la stabilité de l'alliance,

reste également au centre des préoccupations. Elle ne va pas sans poser question à la France, qui n'encourage pas l'examen, sans cesse reporté, des recommandations d'ouverture des négociations d'adhésion. Notre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées reste également très réservée sur la question de l'élargissement européen, lui préférant une refondation au préalable. Pour conclure, l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN constitue une avancée significative pour la stabilité politique de la région et s'inscrit dans une dynamique vertueuse d'intégration.

C'est d'autant plus vrai que la Russie ne cesse de resserrer ses liens avec les peuples slaves, notamment pour éviter que la Serbie et la République serbe de Bosnie n'adhèrent à l'OTAN. On connaît les méthodes de la Russie : le, comme on dit en bon français, qu'il soit médiatique, culturel ou même religieux- je pense notamment aux liens entre les patriarcats de Moscou et de Belgrade ; la « diplomatie Gazprom

la Russie. Le parti de gauche en Macédoine, le Levica, s'oppose fortement à l'adhésion à l'OTAN et dénonce la stratégie des États-Unis, qu'il juge dangereuse pour la paix dans le contexte géopolitique actuel,

Il faut, d'abord, noter que le processus fut long, puisque la Macédoine a adhéré au partenariat pour la paix de l'OTAN dès 1995 et qu'elle participe depuis 1999 au plan d'action pour son adhésion, qu'elle présente, avec raison, comme le gage de son ancrage dans le monde occidental et le symbole d'une reconnaissance internationale à laquelle elle aspire. Il faut aussi reconnaître que, après l'ère autoritaire et clientéliste du gouvernement de Nikola Gruevski, de 2006 à 2016, le gouvernement du Premier ministre

du 12 juin 2018, qui a mis fin à trois décennies de dispute avec la Grèce sur le nom du pays, ainsi qu'avec le traité d'amitié avec la Bulgarie, après soixante-quinze ans de relations conflictuelles entre Skopje et Sofia.

: alors que la déstabilisation s'aggrave en Syrie et devant le manque de fiabilité- c'est le moins que l'on puisse dire -de la Turquie, pourtant membre de l'OTAN, la consolidation de l'architecture de sécurité des Balkans s'impose.

Au regard de ce qui se passe en Syrie depuis quelques jours, on s'interroge sur le rôle de l'organisation. En effet, dans le nord de la Syrie, la Turquie agit non seulement seule, mais au mépris de tous ses engagements à l'égard de ses alliés. Elle semble n'écouter que ce que lui dit la Russie, la Russie, à laquelle, de surcroît, elle vient d'acheter des missiles. L'OTAN est décidément bien malade, et nous n'échapperons pas à une réflexion sur son avenir dans les prochains mois et les prochaines années. Pour autant, le groupe socialiste

depuis sa déclaration d'indépendance en 1991, la République de Macédoine du Nord a souhaité intégrer quelques-unes des grandes organisations internationales pour affirmer d'emblée son identité. Si son entrée à l'ONU a pu se faire dès 1993 sous un nom provisoire, son arrimage à l'OTAN a été compliqué, la Grèce contestant le choix par Skopje du nom de « République de Macédoine Les deux pays avaient, en effet, ouvert un contentieux animé par des enjeux identitaires sur fond d'héritage culturel et patrimonial, un désaccord qui a longtemps brouillé les relations entre la Grèce et la Macédoine. Notre collègue Notre collègue rapporteur, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, l'a rappelé, la recherche d'une solution sur un nom mutuellement acceptable conditionnait l'entrée de la Macédoine du Nord dans l'OTAN, selon le principe affirmé au sommet de Bucarest, en 2008. Je souhaitais souligner que cette posture de prudence, adoptée par les membres de l'organisation, a été la bonne. bonne. Nonobstant l'obstacle du nom, la Macédoine du Nord avait acquis en 1999 le statut de pays candidat à l'alliance atlantique suivi d'un plan d'action pour l'adhésion. La voie était donc ouverte. En ce qui concerne la Grèce, au regard de ses qualités de membre de l'OTAN depuis 1952 et de l'Union européenne depuis 1981, nous lui devions certains égards. Au sein de l'alliance, la Grèce occupe une position stratégique dans la région Sud, à proximité de l'Europe du Sud-Est, de la Méditerranée orientale, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, une zone dont nous connaissons les enjeux stratégiques pour notre sécurité. Cette situation consacre Athènes comme un acteur important de la stabilité de l'Europe.

il a fallu beaucoup de volonté de la part des deux chefs de gouvernement concernés, Zoran Zaev, côté macédonien, et Alexis Tsipras, côté grec, face aux droites nationalistes, lesquelles ont été particulièrement actives dans les deux pays pour tenter de saboter l'accord. Comme l'a rappelé notre collègue rapporteur, au terme des quelques dernières notifications de ratification du protocole d'adhésion signé le 6 février dernier entre l'OTAN et la Macédoine du Nord, cette dernière deviendra le trentième pays membre de l'alliance. Le RDSE approuvera évidemment le projet de loi de ratification du protocole précité. Je mets de côté la très faible contribution financière de la Macédoine du Nord à l'OTAN : on ne peut guère exiger plus de ce pays, compte tenu de son niveau économique.

Néanmoins, je m'attarderai sur la problématique plus générale de l'élargissement sans fin de l'OTAN. On connaît l'impact sur la Russie de la politique dite de la « porte ouverte » vers l'Est, menée par l'organisation. C'est une préoccupation régulièrement exprimée au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.

Lors d'une visite à Belgrade au début de l'année, Vladimir Poutine s'en est pris une nouvelle fois à cette doctrine de l'OTAN, la qualifiant de « vestige de la guerre froide » et de « stratégie militaire et politique mal inspirée et destructrice », qui

la Russie est un acteur incontournable pour la maîtrise des armements conventionnels ou pour résoudre les crises en Syrie, en Iran ou en Ukraine ; l'actualité est là pour nous le rappeler. Enfin, sans entamer un vaste débat aujourd'hui, la réflexion sur les limites de l'élargissement de l'OTAN

On peut certes arguer que la Macédoine du Nord ne remplit pas à ce jour les conditions pour intégrer le marché commun, mais cela finira par arriver. Par conséquent, la question est plutôt de savoir si le fonctionnement actuel de l'Union européenne lui permet de s'élargir encore et encore. C'est la position que la France a exprimée mardi dernier au Luxembourg, en rappelant la nécessité de s'interroger sur les bases de l'élargissement avant d'accepter de nouveaux États membres, et qu'elle a confirmée hier en opposant son veto à la Macédoine du Nord, ainsi qu'à l'Albanie. Sachez, monsieur

Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, madame le rapporteur, mes chers collègues, après l'entrée de la Slovénie en 2004, de la Croatie et de l'Albanie en 2009, et du Monténégro en 2017, la Macédoine du Nord deviendra, si le Sénat approuve ce projet de loi, le cinquième pays des Balkans occidentaux à rejoindre l'alliance atlantique. Disons-le d'emblée : le groupe Les Républicains du Sénat votera en faveur de cette adhésion.

Ce nouvel élargissement s'inscrit réalité dans le droit fil de la politique de la « porte ouverte » de l'OTAN à l'égard des anciens pays du bloc soviétique, après la chute du rideau de fer. Après plusieurs siècles de conflits meurtriers, l'adhésion des pays des Balkans occidentaux à l'OTAN permettra de sceller la réunification du continent européen et sera un gage de paix et de sécurité pour l'Europe. Cet élargissement consacre les efforts importants réalisés par la Macédoine du Nord dans son processus de transition démocratique et sa contribution à la stabilité de la région. je pense au compromis trouvé avec la Grèce sur la question sensible de la dénomination du pays, entériné par l'accord de Prespa du 17 juin 2018, ou à la politique d'apaisement des tensions entre les différentes composantes de sa population. Depuis l'occupation par l'Empire ottoman et les guerres balkaniques jusqu'aux conflits meurtriers de Bosnie-Herzégovine et du Kosovo, nous savons combien cette région a souffert des tensions entre les différentes communautés. Comme le disait Churchill à son propos : « Cet espace produit plus d'histoire qu'il n'en peut consommer ! » L'adhésion de la Macédoine du Nord à l'alliance atlantique aura des répercussions positives sur la région des Balkans, mais elle répond aussi à une cohérence stratégique dont le continent européen a besoin. Cet élargissement de l'OTAN intervient toutefois dans un contexte géopolitique particulier. L'intervention de la Turquie, membre fondateur, au nord de la Syrie contre les combattants kurdes, qui ont été nos alliés contre les groupes terroristes de Daech, pose problème, nous amenant à nous interroger sur l'essence même de l'alliance, sur ses valeurs comme sur la nécessaire communauté d'objectifs. Cette offensive présente un risque majeur de déstabilisation, alors que des centaines de djihadistes étrangers, dont plusieurs Français, sont détenues par les combattants kurdes dans cette zone. considérer la place de la Russie dans l'architecture européenne de sécurité et l'évolution des relations transatlantiques face à la politique unilatéraliste du président américain Donald Trump. Trump. Une réflexion sur l'évolution du rôle de l'OTAN et de l'architecture européenne de sécurité est indispensable. Il est temps de rappeler que l'alliance doit d'abord reposer sur un partage de valeurs, comme le respect des droits humains. L'organisation ne peut fonctionner en « réaction contre une nation ». Monsieur le secrétaire d'État, la France et tous ses alliés doivent prendre des initiatives communes à ce sujet. Permettez-moi sujet. Permettez-moi de conclure mon intervention en évoquant la question de l'élargissement de l'Union européenne, en ma qualité de présidente du groupe d'amitié France-Balkans occidentaux du Sénat. Entendons-nous bien : cette question est tout à fait distincte de l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'OTAN. Notre collègue rapporteur Joëlle Garriaud-Maylam l'a rappelé en commission des affaires étrangères : il n'y a aucune « automaticité Néanmoins, les chefs d'État et de gouvernement devront se prononcer, lors du Conseil européen qui se tient aujourd'hui même, sur la question de l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne avec l'Albanie et la Macédoine du Nord. Or la majorité de nos partenaires européens y sont favorables. Cette adhésion ne représente qu'une étape sur le chemin de l'adhésion de ces pays à l'Union européenne, qui ne serait envisageable qu'à l'issue d'un long processus de plusieurs années et d'une profonde refondation de l'Union européenne après

du processus d'élargissement, avec une plus forte conditionnalité et une nouvelle approche de la négociation par chapitres ? Certes, les pays des Balkans ont encore d'importants efforts à accomplir pour respecter l'ensemble des critères, notamment en matière de lutte contre la corruption, contre les trafics sous toutes leurs formes, contre les mafias qui gangrènent l'économie et pour le respect de l'État de droit. Quelle que soit la décision du Conseil européen, il nous faudra être attentifs à l'aspiration profonde de ces peuples qui frappent depuis plus de vingt ans à notre porte. De la même manière, il nous faudra engager une coopération sur des thèmes majeurs. Ces pays doivent faire face aux crises migratoires et ont besoin d'aide. Pour mémoire, la Macédoine du Nord a dû gérer l'afflux de près de 90 000 personnes en 2016. Rien ne serait plus dangereux que de laisser ces pays se détourner de l'Europe pour se tourner vers d'autres partenaires, comme la Turquie ou la Chine. Nous avons des intérêts à faire valoir, par exemple en ce qui concerne la lutte contre la criminalité et l'immigration clandestine, face au risque d'une nouvelle vague de migrants venant de Turquie. Comme l'a souligné le Président de la République le 29 avril dernier, la France a un rôle important à jouer dans les Balkans. Nous devons renforcer notre place et notre influence dans cette région en matière politique, économique et culturelle, notamment par rapport à nos amis allemands. Très

de certains standards, investir et s'équiper. Il faut que d'autres membres de l'OTAN que les seuls Américains- je pense notamment aux Français

maintenant examiner le début du commencement du processus d'adhésion à l'Union européenne avec un regard quelque peu nouveau et différent. J'en veux pour preuve les accusations dont la France a fait l'objet à l'issue d'un conseil des ministres de l'Europe, laissant à croire que notre pays s'opposerait systématiquement à toutes les nouvelles adhésions. Tel n'est pas le sens de notre démarche. Le Président de la République l'a dit et

la ratification du protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Macédoine du Nord (projet n°

La séance est reprise. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour un rappel au règlement. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce rappel au règlement se fonde sur l'article 36 de notre règlement, qui est relatif à l'organisation de nos débats. Monsieur le ministre, vous avez adressé hier en fin de journée un courrier à l'ensemble des maires

Oui, j'ai signé une tribune, que j'ai postée sur les réseaux sociaux, dans laquelle je réaffirme les orientations du projet de loi que j'ai défendu en conseil des ministres et que j'ai déposé, au nom du Gouvernement, sur le bureau des deux assemblées. Oui, il se trouve que je ne suis pas le directeur général des collectivités locales- je n'en ai ni les capacités ni des moyens-, mais le ministre en charge des collectivités locales. Or le ministre en charge des collectivités locales

Et je pense que le ministre, plus que tout autre, doit être totalement respectueux de ce qu'est la loi et de ce qu'elle n'est pas : tant qu'elle n'est pas adoptée par le Parlement, ce n'est qu'une loi en devenir et en discussion. Acte vous

le ministre est un homme politique, et il a le droit de dire ce qu'il veut. Et les parlementaires sont des hommes ou des femmes politiques, qui ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Je suis sidéré que l'on en soit à dire

peut être reconnu établissement public de gestion et d'aménagement des eaux, c'est-à-dire Épage, et/ou établissement public territorial de bassin,

En outre, les missions des EPTB, telles qu'elles sont définies par l'article 213-12 du code de l'environnement, comprennent l'intégralité des missions des Épage. Dès lors,

la délégation de telles missions à l'ensemble des syndicats de communes ou des syndicats mixtes. Une telle dérogation devait assouplir l'organisation de la compétence « Gemapi » sur les territoires, étant donné que les transformations de syndicats déjà existants en Épage et en EPTB sont parfois longues à être mises en oeuvre. Toutefois, cette échéance du

Les regroupements d'établissements en groupements de coopération sociale et médico-sociale ont permis de réaliser des économies notables, de progresser en termes de qualité d'accueil et d'accompagnement des personnes accueillies et de répondre positivement à toutes les obligations légales. Toutefois, ils trouvent aujourd'hui leurs limites en termes de développement. En effet, ils ne relèvent pas d'une entité juridique unique qui leur permettrait de signer un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens communs. En outre, ils restent fragiles financièrement, avec une capacité d'investissement malheureusement réduite.

dont les Ehpad. Or de tels syndicats pourraient se révéler des outils performants de gestion pour ces établissements, au plus près des besoins des populations et en lien avec les communes qui les composent. Ils permettraient de dépasser les limites des EPCI, donc d'inscrire l'action territoriale dans la réalité des bassins de vie. Afin de favoriser le rapprochement des collectivités territoriales en la matière, je demande un rapport au Gouvernement

Dans l'Hérault, cela concerne plusieurs Ehpad, mais il en existe des dizaines en France, qui se trouvent dans l'illégalité, alors que leurs outils de gestion sont performants, en lien avec les communes et au plus près des populations. Les syndicats permettent de dépasser les limites des communautés de communes et d'inscrire l'action territoriale dans les bassins de vie.

participer financièrement et aider les entreprises concernées. Voilà qui laisse entendre beaucoup de générosité ! Les

Par conséquent, ce n'est pas simplement le montant des dépenses qu'il faut examiner, c'est le principe et, surtout, le fait que l'on met le doigt dans un engrenage, qui entraînera tout le bras, et davantage encore.

cet amendement vise à permettre à un conseil départemental de déléguer à son président l'octroi d'aides dans des circonstances exceptionnelles, lorsque survient une catastrophe naturelle ou un événement

Nouvelles stars du web ou leaders d'opinion des temps modernes, les influenceurs envahissent les réseaux sociaux, au profit de marques qui cherchent à doper leur visibilité et leurs ventes. Cette pratique a tendance à s'étendre aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics et à leurs groupements pour la promotion de leurs actions, de leurs réalisations ou de leur territoire. Il convient de l'encadrer, afin de garantir une plus grande transparence dans les partenariats noués avec des influenceurs, surtout en période préélectorale. Je propose donc de rendre clairement identifiable la personne morale pour le compte de laquelle la promotion est réalisée. avec M. le rapporteur.

le Calvados, arrivent tardivement, trois ans et demi après la création des communes, engendrant un certain nombre de difficultés. En effet, les budgets ont déjà été fondus, les fonctionnaires réunis au sein de la même instance et des subventions attribuées globalement.

que la fusion de deux communes doit faire l'objet d'une « consultation » des administrés des communes concernées. Cette disposition permettrait de renouer le lien entre citoyens et prises de décisions locales. À l'heure où le mouvement de « métropolisation » fragilise de plus en plus les communes et leur pouvoir, il est important de renouer avec plus de proximité, ce qui vaut, aussi, pour la création des différents types d'EPCI. Si commune nouvelle il y a, celle-ci doit s'inscrire dans un projet de territoire commun.

au travers de cet amendement est de nature à renforcer la démocratie de proximité, en obligeant toutes les communes concernées par une fusion à organiser une consultation citoyenne. Cet avis simple et non conforme permettrait à l'assemblée délibérante de connaître l'opinion des administrés, tout en conservant son pouvoir décisionnel.

de la part des élus et de la part des citoyens. Cela permet de mûrir les réflexions. Cela permet à tout un chacun de s'approprier les enjeux. Cela permet de débattre,

de décisions d'élus largement concertées avec la population et qui viennent juste épouser la manière dont les habitants vivent.

impose, à ceux qui souhaitent constituer une commune nouvelle, de l'inscrire dans leur programme électoral. Cela me semble être la base, même si nous ne rendons pas le référendum obligatoire

le rapporteur l'a brillamment rappelé à l'instant. Cela étant, je suis trop attaché à la coopération intercommunale pour ne pas rester

vote. Effectivement, lors de la discussion, au printemps dernier, sur l'organisation des communes nouvelles, nous avions déjà eu ce débat. J'avais personnellement déposé un amendement visant

dissimulé leur volonté de créer une commune nouvelle. Ils ont fait délibérer leurs conseils municipaux, et ceux-ci ont délibéré en ce sens. Quand la population, qui n'avait pas été consultée, a appris le résultat de ces conseils municipaux, il y a eu comme un vent de folie.

de la démocratie ou considéreraient qu'on ne doit pas associer les citoyens aux décisions. M. le ministre a expliqué quels étaient la force et le poids de la démocratie représentative.

cela s'est bien passé. Cette législation avait été demandée et rédigée, avant que nous en débattions, par l'Association des maires de France,

parmi eux des femmes et des hommes pour approfondir les questions et prendre un certain nombre de décisions très importantes pour l'avenir. Ce n'est pas parce que l'on rencontrerait, ici ou là, une difficulté particulière qu'il faut mettre par terre

privées de leurs ressources et de leurs compétences. Elles retrouvent un ballon d'oxygène en s'associant, dans la proximité, avec les communes rurales voisines pour former une commune nouvelle, à plusieurs clochers, mais avec en partage l'école, le service de santé, la résidence pour personnes âgées et les installations sportives que la population des communes membres de la commune nouvelle fréquentait d'ores et déjà, sans pour autant toujours contribuer à la dépense.

soit à l'initiative de ces regroupements. Nous sauvons la vitalité de nos communes rurales et nous leur permettons de compter au sein des grandes intercommunalités Continuons à être favorables au développement des communes nouvelles sur la base de la liberté, sans mettre par terre le système voulu par l'AMF, qui, jusqu'à présent, a bien fonctionné

ce qui peut heurter leur sensibilité. Mais, de grâce, n'hystérisons pas le sujet de façon manichéenne en donnant le sentiment que l'absence de référendum

Le scrutin est clos. J'invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.